La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 18 juin 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

c'est-à-dire des articles 59 à 66 , afin qu'il soit examiné ce soir, à la reprise de nos travaux. Quel est l'avis de la commission

afin que le vélo soit une solution de rabattement vers les gares. Ainsi, nous proposons que les gares ferroviaires et routières, ainsi que les pôles d'échanges multimodaux, soient dotées, d'ici à 2024, d'équipements de stationnement de vélo représentant au moins 6 % du trafic quotidien de voyageurs,

que les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routières doivent s'équiper de parcs de stationnement sécurisés pour les vélos avant le 1 janvier 2024. Par ailleurs, le seuil retenu

des collectivités territoriales, dans la limite de 300 mètres autour des gares du Grand Paris Express. Cette participation minoritaire de la SGP favoriserait l'intermodalité autour des gares

la croissance verte -ont introduit l'obligation d'installer un parc de stationnement sécurisé pour les vélos dans les bâtiments neufs à usage de logement et de bureaux et dans les bâtiments hébergeant un service public industriel, les centres commerciaux et les cinémas neufs. Il convient d'aller encore plus loin et de permettre aux propriétaires ou aux locataires d'un immeuble déjà bâti déjà bâti disposant d'espaces communs suffisants d'installer, à leurs frais, des infrastructures pour le stationnement des vélos. L'article 26 du présent projet de loi prévoit la mise en place d'infrastructures collectives de recharge électrique dans les immeubles collectifs, afin de favoriser le développement des motorisations concernées.

monsieur le ministre copropriétaire. En revanche, le dispositif de la passerelle permet d'ores et déjà de passer de la majorité absolue à une majorité simple, dès lors que la décision a recueilli un minimum d'adhésions des copropriétaires. Le mécanisme de la LOM

L'avantage de ces nouveaux dispositifs est qu'ils sont d'une grande efficacité énergétique ; ils font en outre partie des mobilités actives et contribuent de ce fait à améliorer la santé des personnes qui les utilisent. Aussi cet amendement a-t-il pour objet de demander un rapport

objet de préciser que ces opérateurs et le gestionnaire de réseau doivent présenter l'ensemble des coûts afférents au raccordement, à l'installation et à l'utilisation de la borne de recharge par l'utilisateur. est à M. Bruno Rojouan. Cet amendement vise à contraindre les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique et le gestionnaire du réseau à présenter dans leur devis les délais et les conditions de leur intervention.

Cet amendement vise à favoriser une concurrence saine entre les opérateurs de bornes de recharge et le gestionnaire de réseau, au bénéfice du consommateur, lequel doit être en mesure de faire un choix éclairé.

: La parole est à M. Bruno Rojouan. Le copropriétaire étant le bénéficiaire de la valorisation de son actif immobilier, il lui revient de payer la contribution pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'un des principaux freins au développement de la mobilité électrique et à la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables réside dans la difficulté d'installer des bornes de recharge dans les collectifs. En adoptant l'article 26 , l'Assemblée nationale a pris plusieurs dispositions destinées à faciliter l'installation d'infrastructures de recharge collectives dans les immeubles collectifs existants. Ces mesures vont dans le bon sens, mais elles nécessitent qu'une décision d'équipement soit prise

Il est donc proposé que les immeubles neufs soient livrés, d'emblée, avec une infrastructure électrique commune permettant à chaque occupant détenteur d'un emplacement de stationnement de s'y raccorder. Les coûts correspondants sont minimes au regard de l'avantage de pouvoir ainsi disposer d'un tel emplacement au standard « EV Ready

fait pour la colonne montante de l'immeuble, de la transférer au gestionnaire du réseau de distribution ou de réaliser une infrastructure privée en aval d'un compteur principal dédié et d'en confier la gestion et l'entretien à un opérateur de son choix.

? Si la version initiale de l'article faisait peser une charge trop lourde sur les entreprises disposant de flottes de véhicules, les travaux de notre commission et de la commission des lois ont permis de trouver un meilleur équilibre. Il me paraît nécessaire de conserver des objectifs de renouvellement,

au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues doivent, d'une part, s'assurer qu'une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions déclarer la part de vélos et de véhicules à très faibles émissions. Il conviendrait également d'améliorer l'information des utilisateurs de ces plateformes sur le type de véhicule utilisé

pour assurer leur service.

l'utilisation professionnelle de cycles avec ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque, pour la livraison urbaine, et, plus largement, pour les déplacements professionnels. L'Ademe a validé le référentiel et la définition proposés par l'association Les Boîtes à vélo : le vélo-cargo est défini comme un cycle, à deux ou trois roues, vendu pour transporter le pilote et une charge supérieure à 45 kilogrammes. La logistique urbaine du dernier kilomètre représente un défi considérable pour les territoires urbains et les acteurs Génératrice d'embouteillages- elle représente 20 % du trafic automobile -, d'émissions de gaz à effet de serre- 15 % des émissions de CO2 sont dues au transport de marchandises de pollution de l'air- elle représente 30 % de la pollution en ville -et de nuisances sonores, la logistique est pourtant indispensable au bon fonctionnement des villes. La cyclo-logistique constitue une réponse durable à l'essor de la livraison et aux émissions de gaz à effet de serre qui l'accompagnent. Propre, silencieuse et limitant l'encombrement, elle se substitue avec efficacité aux véhicules utilitaires légers. Intégrer la problématique de la mobilité professionnelle durable dans les plans de mobilité permettra d'anticiper et d'accompagner au mieux le développement des usages.

: il s'agit de la cyclo-logistique. Il y a encore quelques années, ce sujet passait pour un gadget d'écolos rêveurs. Aujourd'hui, tout le monde constate que les vélos-cargos sont de plus en plus présents dans nos villes. À Strasbourg, par exemple, les sacs de farine de l'essentiel des boulangeries du centre-ville arrivent en barge depuis le port autonome jusqu'au bord de l'ellipse insulaire et effectuent leurs derniers kilomètres en cargos-cycles

ainsi explicitement désigné. En effet, si la cyclo-logistique peut être pertinente, son utilité varie grandement selon les entreprises et les environnements.

ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque, pour la livraison urbaine et, plus largement, pour les déplacements professionnels. J'avais déposé un amendement similaire, lequel a malheureusement été frappé du sceau de l'article 40. Je tiens toutefois à réaffirmer mon attachement à ces modes de transport innovants. Nous savons que le dernier kilomètre est le talon d'Achille de la logistique. À Paris, un véhicule sur cinq en circulation livre des marchandises. Or, pour ce fameux dernier kilomètre, les modes massifiés ne peuvent être d'aucune aide : la route est indispensable. Il est toutefois possible de verdir ce dernier kilomètre. À cet égard, l'Assemblée nationale a voté l'extension de la prime à la conversion à l'acquisition d'un vélo-cargo.

Toutefois, la rédaction retenue par nos collègues députés risque de créer de fait une tutelle d'une collectivité sur une autre, en obligeant les autorités organisatrices de la mobilité à intégrer, tels quels, ces schémas dans leurs plans de mobilité.

territoriale (SCoT). Je rappelle que le lien d'opposabilité entre plan de mobilité et schéma de cohérence territoriale existe déjà : c'est le plan de mobilité qui doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale. La création d'un nouveau lien juridique dans le sens inverse

réhabilitant une voie hors agglomération d'y étudier la mise en place d'un aménagement cyclable. En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont à fort trafic, ce qui est rare et peu compatible avec la cohabitation vélos et voitures, mais possible dans des secteurs contraints et généralement en entrée d'agglomération, un aménagement est indispensable. Si ce sont des voies à faible trafic, celui-ci est supposé justifier l'absence d'aménagement dédié aux cyclistes. Pour autant, il n'entraîne pas une réduction des vitesses des rares véhicules utilisant ces voies. Le danger est donc patent et ressenti par de nombreux cyclistes. L'objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement correct ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret et inférieure ou égale à 50 kilomètres

Cependant, le dispositif proposé me paraît aller trop loin, notamment parce qu'il vise à imposer des restrictions de vitesse de circulation à certaines sections de route qui ne seraient pas conformes à certains critères. À cet égard, il me semble plus juste de laisser

véhicules par des emplacements pour vélos sur certains parkings. Pour ce faire, il prévoyait de diminuer le nombre de places de parking lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés permettant un stationnement sécurisé pour au moins six vélos. La commission a considéré que cette disposition était satisfaite

à Mme Colette Mélot. Le développement des mobilités douces, et singulièrement du vélo, repose en grande partie sur l'existence d'infrastructures adaptées à leur stationnement à proximité du domicile des usagers. Le déficit de ces infrastructures constitue aujourd'hui un frein au développement du vélo, notamment tel qu'il est prévu par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Afin d'encourager les mobilités douces, de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter l'artificialisation des sols, il paraît opportun non pas de cumuler les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, mais de mutualiser les surfaces qui doivent y être consacrées. L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme prévoit déjà la réduction d'au moins 15 des aires de stationnement imposées par le règlement du plan local d'urbanisme pour les véhicules motorisés, en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. Le présent amendement vise à compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre d'aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos.

filières. Il participe également à une électrification des usages alors même que d'autres carburants alternatifs participent à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. La création d'un schéma similaire pour la mobilité gaz permettrait de résorber les lacunes du maillage des stations d'avitaillement en GNV en France.

la commission ? La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit que la France doit s'équiper d'un certain nombre de bornes GNV d'ici à 2023 et 2028. Interrogé sur ce sujet, le Gouvernement nous a informés que la trajectoire de déploiement correspondait aux objectifs fixés et que les besoins en planification et développement n'étaient pas de la même envergure que pour l'électromobilité. Néanmoins, je suis sensible aux besoins de donner à la filière toutes les garanties et d'assurer le pilotage de l'offre en GNV afin qu'elle corresponde aux besoins du

une planification partagée des infrastructures de recharge qui ne se limite pas au GNV et à l'électrique, mais s'étende aux biocarburants et à l'hydrogène. Mon ministère va lancer dans les prochains jours, au sein de la pour la transition énergétique du transport routier

Les ZFE sont un important levier de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de l'air dans les zones les plus denses. Il n'en demeure pas moins que leur mise en place, qui passe par des restrictions de circulation des catégories de véhicules les plus polluants, est susceptible de susciter de l'incompréhension, voire des crispations, chez nos concitoyens.

La commission a donc proposé plusieurs évolutions concernant les ZFE rendues obligatoires par la LOM et qui connaîtraient encore des dépassements des seuils de qualité de l'air. En lien avec le rapporteur pour avis de la commission des lois, assoupli les schémas de restriction de circulation sur deux points : d'une part, en redonnant la main aux collectivités territoriales pour la définition de leur schéma de restriction de circulation

On peut comprendre que les constructeurs automobiles soient favorables aux ZFE, car elles vont permettre de moderniser le parc automobile- dont acte -, mais pensons à ceux qui n'auront pas les moyens

mobilité (ZFE-m) dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Je comprends l'impératif de lutter contre la pollution de l'air et de mettre en place des zones à faibles émissions.

au sein des ZFE, à limiter cette dérogation aux déplacements non professionnels afin d'éviter tout effet d'aubaine et à porter de 30 à 40 ans l'âge minimal d'entrée en collection, toujours afin d'éviter tout effet d'aubaine. La parole

Ces dernières années, la France a régulièrement été rappelée à l'ordre par Bruxelles pour non-respect des normes européennes sur les concentrations dans l'air en oxyde d'azote et en particules fines PM10. En l'absence de vent, ces seuils sont régulièrement dépassés dans plusieurs agglomérations françaises. Pour parvenir à faire baisser la pollution atmosphérique, le Gouvernement cible le trafic routier, responsable de 30 % des émissions directes de particules fines et de 60 % des émissions d'oxyde d'azote.

agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici au 31 décembre 2024. Il prévoit également d'imposer un schéma de restriction progressive de la circulation des véhicules les plus polluants en vue d'une interdiction définitive dans les ZFE-m en 2025. Il apparaît aujourd'hui indispensable de déployer les ZFE-m le plus largement possible, selon un calendrier réaliste, mais néanmoins ambitieux.

de mettre en place des zones à faibles émissions mobilité aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants et aux véhicules utilitaires légers d'ici au 31 décembre 2024, qui n'a fait

La mesure signerait, par exemple, la disparition des marchés non sédentaires dans les zones concernées. Il conviendrait, à tout le moins, que la mise en place des ZFE tienne compte non seulement de l'offre existante de véhicules propres

De même, l'obligation d'affichage de l'impact environnemental des produits et services est prématurée dans la mesure où l'expérimentation en cours n'a même pas fait l'objet d'un bilan. Il serait logique et cohérent qu'une telle mesure, qui va nécessairement peser sur les entreprises, notamment sur les plus petites d'entre elles, soit prise à l'échelle de l'Union européenne, ne serait-ce que pour déterminer une méthodologie commune- là encore, il s'agit d'une simple question de bon sens Il faut certes décarboner l'économie française, mais cela ne peut se faire qu'avec un accompagnement des acteurs économiques, notamment des PME et des TPE.

Ce projet de loi prévoit d'aller plus avant en étendant la mise en place des ZFE aux agglomérations de plus de 150 000 habitants. Les ZFE ne sont pas une lubie d'écologistes maximalistes : c'est une démarche européenne déjà mise en place dans plus de 200 villes, qui restreignent l'usage des véhicules les plus polluants. Restreindre l'usage de véhicules polluants tout en maintenant le droit au déplacement et en tenant compte des réalités disparates des territoires, des activités sociales et économiques : l'enjeu est complexe. Et les inquiétudes, les mécontentements, les crispations ne viseront d'abord ni l'Europe, ni l'État, ni même nous, parlementaires, mais principalement les élus locaux.

de laisser aux alternatives le temps de se développer. Je tiens aussi à saluer la mise en place de mesures incitatives comme la création d'un prêt à taux zéro pour accompagner les ménages les plus précaires dans le renouvellement de leur véhicule. Je salue également le fait de redonner de la souplesse aux maires en leur permettant de conserver leur

par exemple, le souhait d'interdire les véhicules Crit'Air 2 au 1 janvier 2028 suscite de vives et légitimes inquiétudes et oppositions. Comment imaginer qu'en 2028, c'est-à-dire demain, près de 180 000 véhicules immatriculés du parc automobile actuel ne pourront plus rouler dans aucune

Agir de manière précipitée et pénalisante serait particulièrement contre-productif, voire dangereux. Grâce au travail sénatorial,

les personnes souhaitant effectuer cette transition énergétique. Néanmoins, les collectivités seront libres de mettre en place les schémas de restriction de circulation qu'elles souhaiteront, sur le périmètre de leur choix, et selon un calendrier qui pourra être progressif.

les critères permettant d'établir que l'obligation de mettre en place une ZFE est satisfaite sur un territoire donné. L'Assemblée nationale avait précisé qu'une ZFE est considérée comme mise en place si elle couvre la majeure partie du territoire.

pourrait donc aboutir à la création de ZFE très vastes, donc plus coûteuses et difficiles à contrôler, qui ne produiraient pas l'effet voulu sur la santé et l'environnement des habitants concernés. Il me paraît donc plus pertinent de retenir le critère de « majeure partie de la population ». Une telle précision assurera la cohérence entre le périmètre des ZFE et les besoins en termes de qualité de l'air.

serait comprise, je le crains, comme une incitation à reporter toute action déterminante aux prochains mandats municipaux et nous exposerait à des sanctions européennes pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air. La parole est à M. Joël l'amendement n° 1499. Cet article étend, à compter du 31 décembre 2024, l'obligation de création d'une zone à faibles émissions mobilité aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Il précise également, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, les restrictions de circulation à mettre en oeuvre lorsque les seuils de qualité de l'air sont dépassés dans les ZFE rendues obligatoires par la LOM, en fixant le calendrier qui permettra d'atteindre les objectifs de qualité de l'air que la France s'est fixés. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assouplir fortement ce calendrier de restriction de circulation dans Les ZFE-m, en supprimant les étapes intermédiaires. part, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de maintenir ces différentes étapes, au risque de ne pas être en mesure d'atteindre, en 2030, les objectifs fixés en termes de qualité de l'air dans les ZFE-m. L'amendement n° 1972

mobilité en prévoyant le transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m au président de l'EPCI à fiscalité propre, grâce à la création d'un pouvoir de police spéciale. Cette disposition soulève deux difficultés : la première tient à la confusion entre la compétence ZFE-m et le pouvoir de police spéciale ; la seconde, à l'absence

premièrement, de clarifier le dispositif en précisant qu'il s'agit bien d'un transfert des pouvoirs de police spéciale relevant à ce titre de l'article L. 5211-9-2 du code des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, mais aussi de la compétence communale d'instituer volontairement une telle ZFE-m - en dehors des cas obligatoires -, laquelle obéit à des règles de transfert dans le cadre du droit commun. de soumettre cette décision à l'accord du président de l'intercommunalité et des maires des communes concernées par arrêté, à la majorité qualifiée, soit par la moitié au moins des maires de communes regroupant les deux tiers de la population totale de l'EPCI, soit par les deux tiers au moins des maires des communes regroupant 50 % de la population totale. Tel est l'objet de cet amendement, qui permettra une mise en oeuvre rapide et efficiente des ZFE-m. Cet article prévoyait, dans son alinéa 17, un transfert automatique des compétences et prérogatives des maires en matière de ZFE-m au président de l'EPCI. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant un mécanisme visant à empêcher le transfert automatique intercommunale si un tiers des maires ou les maires représentant au moins un tiers de la population de l'établissement ou du groupement s'y opposent. Les auteurs de l'amendement ne sont pas favorables à cette disposition, qui permet de mettre fin au transfert de compétences pour toutes les communes concernées.

revenir sur l'équilibre trouvé par la commission. Nous avons en effet considéré que le transfert automatique des pouvoirs de police de ZFE-m des maires aux présidents d'EPCI pourrait nourrir des crispations sur la mise en place des ZFE-m et constituer une atteinte disproportionnée au principe de libre administration des collectivités territoriales. Je suis donc défavorable aux amendements n 2162 et 1501, qui visent à supprimer ce mécanisme.

dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. En revanche, je suis défavorable au reste de l'amendement, qui vise à revenir sur les apports de la commission et à rétablir les schémas de restriction de circulation.

qui a souhaité assouplir le schéma de restriction de circulation dans les ZFE-m rendues obligatoires par la LOM et qui ne respecteraient pas les normes de qualité de l'air. L'idée est de définir un objectif réaliste.

que toutes les ZFE-m prévues n'ont pas été mises en place et que les moyens de contrôle ne sont pas au rendez-vous. Permettez-moi d'apporter une précision sur ce point. Nous avons discuté avec les présidents d'EPCI qui ont mis en place ou essayé de mettre en place des ZFE. Certaines

à discriminer les gens en fonction de leur métier ou de leur capacité à changer plus ou moins vite de véhicule. J'entends déjà, dans la grande banlieue parisienne,

les calendriers retenus ne permettent pas à des milliers de professionnels d'acquérir un véhicule aux normes. Ils se trouvent alors empêchés d'exercer leur métier. Certains des calendriers de restrictions envisagés par les collectivités vont en effet largement au-delà du calendrier proposé dans le projet de loi et prévoient des interdictions de circulation des véhicules classés Crit'Air 2 à compter du 1janvier 2024. Les aides proposées pour le renouvellement du parc de véhicules se révèlent insuffisantes pour certaines catégories de ménages, qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf ou qui doivent, en plus, subir une décote importante de leur ancien véhicule sur le marché de l'occasion du fait de ces futures restrictions Il en sera de même pour de nombreux professionnels, qui n'auront pas pu amortir l'achat de leurs anciens véhicules. Les calendriers des restrictions de circulation décidés par certaines collectivités territoriales auront donc un impact sur la circulation des véhicules des entreprises, des salariés, mais aussi des consommateurs. consommateurs. Au-delà des effets sanitaires et environnementaux, il convient donc de faire en sorte que l'étude réalisée préalablement à l'instauration d'une ZFE-m par les collectivités locales et jointe à l'arrêté soumis à consultation publique, conformément à ce que prévoit la LOM, présente également les impacts socio-économiques du dispositif mis en oeuvre. Cette étude permettrait d'appréhender les enjeux socio-économiques du territoire concerné, de mieux accompagner les acteurs impactés, tels que les professionnels de l'automobile, et d'assurer une plus grande acceptabilité de la population concernée par le dispositif, tout en calibrant au mieux l'accompagnement nécessaire. Quel est l'avis de la commission ? S'il

L'article 27 du présent projet de loi étend l'obligation de créer une zone à faibles émissions mobilité aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants.

de ces véhicules historiques ne permettrait pas d'améliorer de façon significative la qualité de l'air et mettrait à mal un patrimoine culturel vivant, une filière économique représentant 24 000 emplois et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le Le législateur a mis en place les ZFE-m pour lutter contre la pollution due aux véhicules de transport de personnes et de marchandises, mais pas des véhicules ayant une dimension sanitaire, historique, sécuritaire, etc. Cet amendement vise donc donc à prendre en compte au sein des ZFE le cas des véhicules dont l'usage ne se limite pas au transport de personnes et de marchandises, en prévoyant une exception aux restrictions de circulation pour les véhicules de collection. Quel est l'avis de la commission ? Ces dispositions de la commission ? Ces dispositions ne semblent pas nécessaires dans la mesure où, en ce qui concerne les véhicules d'intérêt général, les dérogations aux restrictions de circulation au sein des ZFE sont déjà prévues dans le décret

Par ailleurs, cette mesure est d'ordre réglementaire. Nous avons engagé un travail avec la Fédération française des véhicules d'époque, ainsi qu'avec l'Amicale parlementaire des amis des véhicules de collection. Les prochaines réunions sont prévues en juillet. Je propose de nous en remettre à ce travail et je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur. Monsieur Moga, l'amendement

que le monde des collectionneurs de voitures anciennes est composé de gens passionnés et passionnants, intéressants et désintéressés. Ils sont un maillon essentiel pour faire vivre notre patrimoine,

les rejets de particules de plus de 1 000 tonnes et les rejets de particules d'oxyde d'azote d'environ 25 000 tonnes. Au total, le véhicule ne pollue pas plus qu'en sortie d'usine. La ZFE n'est bien entendu pas remise en cause. Il s'agit de prendre en compte l'effet social d'une mesure qui aboutirait à interdire à des millions de Français l'accès aux agglomérations de plus de 150 000 habitants et conduirait à une ségrégation géographique. Il faut donc laisser les automobilistes qui entretiennent bien leur véhicule, notamment sur la base de cet éco-entretien,

il semble difficile à mettre en oeuvre puisqu'il conduirait à créer un dispositif très complexe : en plus de la vignette Crit'Air, il faudrait se doter d'un nouveau signe distinctif relatif à l'état de santé du véhicule. Deuxièmement, il est susceptible de réduire l'objectif même d'une ZFE puisqu'un véhicule peut être au maximum de ses capacités

Ainsi, une norme applicable à un véhicule Euro 4, même bien entretenu, est nettement supérieure à celles qui sont applicables à un véhicule de norme Euro 6. Pour ces raisons, auxquelles s'ajoutent des motifs de complexité opérationnelle, nous demandons le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Les professionnels ne sont pas opposés à ces exigences, bien au contraire, à condition qu'on leur donne les moyens concrets de continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions et surtout à un coût soutenable, notamment lorsqu'ils parcourent de longues distances en une seule journée. tenu de l'autonomie plus limitée d'un véhicule électrique, du temps de recharge, du nombre insuffisant de bornes de recharge ou de l'absence de ces dernières, ce type de véhicule n'est pas toujours le plus adapté pour bon nombre d'entreprises. Des véhicules fonctionnant avec d'autres technologies, telles que le bioGNV ou l'hydrogène, pourraient, en l'occurrence, être plus adaptés. Après son passage en commission, l'article 27 du projet de loi prévoit que, dans les ZFE-m, « l'autorité compétente s'assure du déploiement et de l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Le présent amendement tend à étendre cette disposition à l'ensemble des véhicules propres, afin de ne pas se cantonner aux seuls véhicules électriques, et à répondre ainsi aux besoins exprimés par les professionnels. Quel de la commission ? L'élargissement des technologies concernées par le déploiement et l'installation d'infrastructures de recharge dans les ZFE-m à l'hydrogène ou au bioGNV semble bienvenu. Je ne dispose néanmoins pas d'assez d'éléments pour évaluer l'impact potentiel de cette précision sur les infrastructures de recharge et ses effets pour les collectivités. C'est la raison pour laquelle je m'en remettrai à l'avis du Gouvernement.

planification concertée, organisée, sur l'ensemble des carburants alternatifs et des énergies- je pense évidemment à l'électrique, à l'hydrogène, au biocarburant, au GNV. Ce travail permettra d'aboutir à l'objectif visé. Je vous demande donc, monsieur le sénateur,

seulement limiter la mobilité des personnes. La mise en place d'une trajectoire pour réduire la pollution liée au transport de marchandises est bien sûr nécessaire.

permettant de faire évoluer la logistique dans les ZFE en réduisant ses émissions et ses nuisances et en l'insérant mieux, notamment par la cyclo-logistique, dans une ville apaisée et respirable. Quel est l'avis de la commission ? Cet

des seuils de répartition des modes de transport. Il me semble que ce n'est pas le rôle d'un président d'EPCI ou d'un maire. De plus, les ZFE-m ont déjà la main en matière de restrictions de circulation. En second lieu, il tend à traiter de manière différenciée les entreprises qui sont volontaires et les autres, mais aussi les entreprises locales et les autres, ce qui conduira à complexifier les modalités de contrôle. L'avis est donc défavorable.

constitue un frein majeur à l'investissement des entreprises et au renouvellement de l'ensemble du parc automobile. Dans les métropoles et les grandes villes, le manque de foncier disponible pour permettre l'installation de ces points d'avitaillement est un sujet de préoccupation majeur pour les professionnels du transport et de la logistique, qui doivent pouvoir s'appuyer sur un maillage suffisant de points d'avitaillement afin d'effectuer leurs tournées. L'État doit favoriser le déploiement de ces infrastructures de manière coordonnée et cohérente. Le présent amendement vise à confier à l'Ademe, organisme que l'on souhaite voir renforcé, la charge de la coordination nationale du développement des nouveaux réseaux de recharge et d'avitaillement nécessaires au soutien du déploiement de technologies propres et économes dans le secteur des transports. Cette mesure lui permettra d'appuyer les communes au moment de la mise en oeuvre des schémas directeurs d'infrastructures de recharge. Quel est l'avis de la commission ? Je suis est l'avis de la commission ? Je suis globalement favorable aux dispositions permettant de renforcer la gouvernance et la prospective en matière de réseaux de recharge. Je m'interroge simplement sur l'articulation envisagée entre les schémas directeurs d'installation des infrastructures de recharge électrique et le rôle de coordination qui serait ainsi confié à l'Ademe.

commission ? Le freinage est une source importante de pollution de l'air, comme vous le savez, mon cher collègue. C'est d'ailleurs l'un des constats formulés par la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux à laquelle nous avons été un certain nombre à participer. En revanche, sur la forme, je m'interroge sur le besoin de préciser par décret les modalités d'équipement des véhicules en matière de freins. Cette mesure pourrait peut-être porter atteinte au principe de neutralité technologique.

10 à 12 du rapport de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. Il émane des deux rapporteurs Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau. Il tend à prévoir un recensement des principaux itinéraires de fuite par arrêté des ministères chargés des transports et de l'intérieur, qui doit être actualisé tous les cinq ans ; une obligation pour le représentant de l'État dans le département dans ces zones de réunir l'ensemble des parties prenantes afin de définir

? Comme le président Longeot, je salue l'excellent travail réalisé par la mission Pointereau-Bonnefoy sur le transport de marchandises.

d'ici au 1 janvier 2023. Ce n'est qu'en cas d'échec des concertations que pourraient être mises en place des zones de réduction des nuisances, cet outil permettant aux maires de protéger leurs communes trop souvent frappées par des reports de trafic pour éviter de payer

oubliées de nos politiques publiques. J'émets donc un avis favorable de nombreux mois. Je précise que le code général des collectivités territoriales permet déjà aux maires de prendre des mesures restreignant ou interdisant l'accès de certaines routes à certains usagers, afin de limiter les nuisances environnementales. De telles mesures sont évidemment

de mettre en oeuvre des ZFE-m et les difficultés qu'elles peuvent susciter. Nous avions trouvé un équilibre en commission sur leur périmètre et sur leur évolution. Il ne me semble pas nécessaire de le modifier avec un nouveau dispositif,

sur les dispositifs « angle mort » des poids lourds. Dans ma vie de cycliste, mes plus grandes frayeurs ont été provoquées par des camions, des camionnettes ou des bus qui ne m'avaient pas vu, car j'étais dans l'angle mort au moment où ils tournaient ou se rabattaient. Dans les ronds-points si mal adaptés au partage entre véhicules motorisés et vélos, ce type de situation est particulièrement fréquent. Je peux dire, en tant que professeur chargé des épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, que les échanges d'expériences avec mes élèves m'ont toujours confirmé que c'était l'un des principaux problèmes. Les chiffres macabres en attestent : à Paris, la moitié des accidents mortels de cyclistes sont liés à une collision avec un poids lourd. Comme les ceintures de sécurité en leur temps ont sauvé des vies, les dispositifs techniques capables de détecter la présence d'un usager vulnérable en sauveront aussi. Ils ne seront obligatoires qu'en 2024 pour les nouveaux véhicules. Cet amendement vise à accélérer leur mise en oeuvre, en premier

la circulation des poids lourds dépourvus d'un dispositif de détection des usagers vulnérables, comme cela a été rappelé à l'instant. Une telle mesure permettrait d'inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d'un dispositif de détection.

d'intégrer des dispositifs techniques permettant d'alerter le conducteur d'un poids lourd de la présence d'un usager vulnérable dans l'un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concernera cependant que les véhicules neufs. Nous proposons d'accélérer cette mise en oeuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase pour la sécurité de tous les usagers de la route. Il s'agit d'inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d'un tel dispositif de détection, tout en laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire. Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d'un urbanisme apaisé, où l'espace public favorise le développement des mobilités actives.

moi aussi qu'il faut renforcer l'attractivité du vélo. Néanmoins, le dispositif proposé ne me semble pas adapté, ces restrictions me paraissant extrêmement difficiles à contrôler sur le terrain. Par ailleurs, et vous l'avez très bien dit, madame Filleul, les maires disposent déjà de pouvoirs de police de circulation qui leur permettent de restreindre le passage de certaines catégories de véhicules. En outre, je suis plus favorable à des mécanismes d'incitation- mise en place de pistes sécurisées, création de bonus pour l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité, comme le prévoit l'article 25 -qu'à une interdiction de circulation pure et simple. Enfin, vous l'avez également rappelé, madame Filleul, le droit européen prévoit que les camions neufs devront être équipés de tels dispositifs au plus tard à compter de 2024,

n'étant pas requis pour ces véhicules individuels, une augmentation du nombre d'accidents est à craindre. Nous le constatons tous les jours, de nombreux usagers méconnaissent les règles élémentaires de prudence. C'est pourquoi il est proposé de compléter l'article 27 AA, introduit au Sénat en commission afin de sensibiliser les futurs usagers de la route aux règles essentielles du code de la route,

le schéma directeur des itinéraires cyclables. Ce document, intégré au plan de mobilité, fait l'objet d'une concertation avec les associations et les habitants ; il permet de donner au vélo toute sa place dans la stratégie de mobilité globale du territoire.

L'article 27 A va plus loin en ce qu'il considère que le besoin est réputé avéré pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une ZFE-m, ainsi que de celles qui desservent ces zones, lorsqu'elles sont situées à moins de cinq kilomètres et sur le territoire de l'EPCI ayant mis en place la ZFE-m. De ce fait, la référence aux orientations en matière de déplacements cyclables, adoptées par les élus locaux dans le cadre des plans de mobilité, disparaîtrait. Or une telle obligation pourrait ne pas correspondre aux besoins locaux. Le présent amendement vise plutôt à prévoir que le besoin est réputé avéré lorsque les aménagements ou itinéraires cyclables sont inscrits dans le schéma directeur des itinéraires cyclables qui est intégré au plan de mobilité. Il tend donc à introduire plus de souplesse pour les collectivités territoriales.

l'obligation de réaliser des aménagements cyclables afin d'offrir aux habitants une alternative au trafic automobile. En revanche, cette obligation ne s'appliquerait pas de manière systématique, elle dépendrait du schéma directeur des itinéraires cyclables.

peu opportunes de réaliser des pistes cyclables sur l'unique fondement de la proximité d'une ZFE-m. De plus, une collectivité pourrait être amenée à renoncer à des travaux de maintenance

proportionnée dans la mesure où l'obligation de réaliser une piste cyclable tombe en cas d'impossibilité technique ou financière justifiée. Le Gouvernement est donc défavorable

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que les informations environnementales devaient notamment concerner les émissions de gaz à effet de serre et à obliger les services numériques d'assistance aux déplacements à à proposer aux utilisateurs un classement des différents itinéraires suggérés selon leur impact environnemental. Nous estimons utile d'inscrire cette précision à l'alinéa 5, et non à l'alinéa 2,

de 2024 afin d'encourager les mobilités partagées, de favoriser des déplacements moins polluants, de contribuer à la transformation des habitudes et d'encourager la pratique du covoiturage sur des distances courtes et moyennes, et plus généralement les mobilités partagées. Cet amendement a été travaillé avec Ecov.

qu'il ne suffit pas de prendre des mesures de restriction de la circulation automobile si, dans le même temps, nous ne créons pas les conditions tarifaires permettant une plus grande utilisation des transports collectifs.

et Île-de-France Mobilités de mettre en place des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs

commission, en accord avec la commission des lois, a estimé que l'obligation d'adopter des barèmes tarifaires favorables aux transports collectifs et favorisant l'intermodalité était non seulement déjà satisfaite- je viens de le dire -, mais qu'elle conduirait surtout à restreindre la liberté tarifaire des régions. C'est la raison pour laquelle la

Ces véhicules électriques partagés répondent parfaitement aux objectifs énoncés dans le code général des collectivités territoriales en matière de redevance de stationnement des véhicules sur voirie, lequel prévoit que le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules et l'utilisation de moyens de transport respectueux de l'environnement. l'aménagement (Cerema) dans une étude de février 2021, le barème tarifaire fixé par l'autorité compétente doit tenir compte de la situation particulière des usagers des véhicules à très faibles émissions mis à leur disposition par les opérateurs de services de partage.

de la commission ? La possibilité de moduler la redevance de stationnement en fonction de l'impact environnemental du véhicule est déjà possible en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Faire de cette possibilité une obligation ne me semble pas nécessaire à ce stade, d'autant moins qu'un certain nombre de villes se sont déjà saisies de cette possibilité. C'est la raison pour laquelle je demande

des villes comme Paris, Nice ou Aix-en-Provence, qui accordent la gratuité de stationnement aux véhicules électriques, qu'ils soient partagés ou non d'ailleurs. Cet amendement étant satisfait, j'en demande le retrait.

L'intermodalité est bénéfique écologiquement, car elle permet de généraliser les transports en commun sur les longs trajets et favorise ainsi les mobilités propres. Elle doit donc être facilitée, notamment par la création d'une carte multimodale. Quel est l'avis de la commission ? La multiplication

semble donc opportun dans la mesure où cela reste un objectif et ne porte pas atteinte à la liberté tarifaire des régions. Je rappelle que plusieurs régions ont déjà mis en place des titres de transport uniques- là non plus, elles n'ont pas attendu la Convention citoyenne

dans le bassin de mobilité. J'ajoute qu'un programme de certificats d'économie d'énergie (C2E) de plusieurs millions d'euros a été lancé récemment, dans le but de développer des interfaces standardisées permettant la création de cartes multimodales. L'amendement étant satisfait, je vous en propose le retrait. Je

qui n'est pas toujours, tant s'en faut, à la hauteur de leurs attentes, notamment en matière de mouvements régionaux pendulaires. C'est particulièrement le cas avec les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Nous prévoyons donc la création d'une modulation des subventions d'exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité, ainsi que d'un mécanisme de baisse des tarifs des abonnements des usagers si la qualité de service est défaillante. Je rappelle que, en 2019, seulement 81,2 % des TER programmés sont arrivés à l'heure ; 9,7 % n'ont pas circulé, et 9,1 % sont arrivés avec un retard supérieur à 5 minutes. Ces résultats, qui ne montrent aucun progrès notable depuis une dizaine d'années, doivent être améliorés, alors même que le télétravail se réduit pour un retour progressif, mais constant des Français vers leur lieu de travail. Quel est l'avis de la commission ? Vous l'avez rappelé,

La création d'un mécanisme de réduction des abonnements en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l'AOM en matière de régularité est donc tout à fait bienvenue. La Cour des comptes, dans son récent rapport sur les TER à l'heure de l'ouverture à la concurrence, reconnaît la nécessité d'accroître l'exigence sur le niveau

dans l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Les Si le droit en vigueur permet le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transports en commun, en réalité, ce cumul n'existe pas. Pourquoi ? À cause du plafond fiscal, fixé à 500 euros par an et par salarié, salarié, alors qu'en Île-de-France le pass Navigo coûte entre 717 euros et 827 euros. Par le présent amendement, nous proposons donc d'exclure le montant annuel de la participation de l'employeur à l'abonnement de transports en commun du calcul de l'avantage fiscal. visons ainsi à favoriser l'intermodalité et la cohésion des territoires, en permettant de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare.

Le forfait mobilités durables est un levier important des politiques de report modal. Dans le secteur privé, il est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transports en commun, mais l'avantage fiscal

le plafond de l'avantage fiscal fixé à 500 euros semble insuffisant et couvre tout juste l'abonnement aux transports en commun. Cet amendement vise donc, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l'abonnement de transports publics, à augmenter ce plafond de 500 euros à 600 euros par an et par salarié.

n° 979 rectifié . Cet amendement vise à généraliser le forfait mobilités durables dans les entreprises de plus de 11 salariés de façon progressive.

. Contrairement au secteur privé associatif et à la fonction publique territoriale, pour lesquels le forfait mobilités durables revêt un caractère facultatif, dans le reste du secteur public- fonction publique hospitalière et d'État -, il est obligatoire. Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés et les fonctionnaires, il est nécessaire de généraliser le dispositif. Tel est l'objet de cet amendement.

et d'ajouter l'application de ce forfait à la fonction publique territoriale à compter du 1 janvier 2024, afin, notamment, de porter de 200 euros à 500 euros le montant de la prise en charge des frais de déplacement par l'employeur.

et 725 rectifié visent à rendre le forfait mobilités durables obligatoire. Au regard des résultats du baromètre « forfait mobilités durables », publié en avril dernier, il apparaît prématuré de recourir à une obligation pure et simple. Il me semble plus opportun de laisser les entreprises s'emparer de ce dispositif dans les conditions fixées au sein des accords d'entreprise ou de branche. Les amendements n 549 rectifié, 597 visent à renforcer les possibilités de cumul entre le forfait mobilités durables et l'abonnement aux transports en commun. Je partage cette préoccupation, mais la solution proposée ne semble pas opérante,

2020. À ce stade, nous ne disposons pas encore de retours suffisants pour préconiser un caractère obligatoire. Nous avons lancé un baromètre, qui monte néanmoins une bonne appropriation du dispositif. Nous avons confié une mission à l'Ademe pour évaluer les mesures collectives et les négociations

d'abord parce qu'ils constituent une dépense obligée pour les ménages populaires ; ensuite parce que leur usage massif est totalement nécessaire face à l'urgence climatique pour décarboner les déplacements du quotidien en réduisant fortement la pratique de l'autosolisme. Le Sénat propose, comme la Convention citoyenne pour le climat, d'abaisser le taux de TVA sur les billets de train à 5,5 %. part, nous proposons d'élargir cette logique à l'ensemble des transports collectifs du quotidien. Cet amendement fait écho à la récente décision allemande d'abaisser le taux de TVA sur les transports collectifs terrestres dans le cadre de son plan climat.

mais la commission a vraiment souhaité envoyer un signal fort à destination du transport ferroviaire en particulier, comme M. le sénateur Laménie L'objectif est notamment d'enclencher la logique du report modal entre le train et l'avion, dont l'écart de prix des billets peut parfois être en décalage avec leurs impacts environnementaux respectifs.

que le transport ferroviaire puisse retrouver, après cette pandémie, des taux de fréquentation suffisamment importants. Nous serons là pour rappeler les opérateurs à leurs obligations tarifaires.

à des prix tout à fait attractifs, non seulement pour les familles, mais aussi pour les usagers individuels. Par ailleurs, en ce qui concerne la TVA, je me dois de dire que, en toute logique budgétaire, il faudrait une équité de traitement pour la partie des transports ferroviaires qui est

qui a été rappelée à l'instant, de la baisse de la TVA dans la restauration, car l'objet n'est pas le même. Cette mesure visait la création d'emplois essentiellement. Là, nous souhaitons respecter le principe « pollueur-payeur

abaisser le taux de TVA à 5,5 % sur les billets de train pour le transport de voyageurs. Bien évidemment, nous nous en félicitons, mais nous considérons néanmoins qu'il est nécessaire d'étendre cette mesure à l'ensemble des transports publics collectifs de personnes, y compris routiers

Ils le déplorent, car ces deux modes de transport participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le transport, avec 33 % des émissions, est le secteur le plus concerné par la nécessaire transition énergétique.

Une réduction du taux de TVA imputée sur le transport fluvial de marchandises à 5,5 % engagerait une diminution des prix favorisant ainsi ce mode de transport. Le présent amendement vise à traduire l'objectif de la Convention citoyenne pour le climat intitulé « Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances, en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial

30 prévoit la définition, tous les cinq ans, d'une stratégie de développement du transport intérieur par les modes massifiés, évaluée chaque année et suivie par des indicateurs précis. Enfin, nous visons, ensemble, l'objectif de doublement de la part

Jean-Pierre Corbisez. Le renouvellement des concessions autoroutières peut constituer l'occasion d'inciter nos concitoyens à recourir au covoiturage et aux transports collectifs, par l'adoption d'une tarification préférentielle des péages pour ces modes de transport. salue, d'abord, l'adoption de cet article en commission. Mais afin d'aller plus loin, nous vous proposons de prévoir, par cet amendement, la mise en place de voies de péage réservées au covoiturage et aux transports collectifs. Disant cela, je ne fais que reprendre la proposition 29 du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières, qui nous a été remis le 16 septembre de l'année dernière. Quel

: La parole est à Mme Angèle Préville. Le présent amendement vise à alerter le Gouvernement sur l'absolue nécessité de revoir les contrats de concession, lorsqu'ils arriveront à échéance, afin de mieux prendre en compte les nouveaux usages de la route, d'introduire de la justice sociale dans le paiement des péages et d'inciter les automobilistes à utiliser les transports alternatifs aux véhicules thermiques individuels, et donc d'inscrire ces infrastructures essentielles essentielles dans la transition écologique. Ainsi, dans l'hypothèse où l'État serait amené à renouveler ces contrats de concession, il apparaît indispensable d'envoyer dès maintenant un message très fort aux sociétés concessionnaires sur l'hypothèse d'un renouvellement ou d'une renégociation de ces contrats. Il s'agirait d'imposer de l'innovation et la présence de services correspondants aux nouveaux usages de la route, notamment le covoiturage. Les émissions de gaz à effet de serre étant étant particulièrement corrélées aux embouteillages, une tarification des péages différenciée pour les heures creuses serait en mesure d'inciter les trafics non contraints à décaler leur passage, assurant ainsi plus de fluidité pour les usagers qui n'ont pas d'autre choix. Cette mesure en faveur de la réduction des gaz à effet de serre devra, par ailleurs, nécessairement s'accompagner de mesures d'accompagnement social des personnes précaires assignées à l'utilisation de leur voiture individuelle pour leurs trajets du quotidien, afin de les aider à changer la motorisation de leur véhicule. Ces dispositions sont d'ores et déjà défendues par les sénateurs socialistes d'autres amendements. La nécessaire transition écologique ne peut se faire sans mesures sociales fortes. de la commission ? La prise en compte, lors du renouvellement des concessions, de mesures participant à décarboner le transport est en effet essentielle. Pour autant, les éléments listés dans cet amendement comme devant être inscrits dans le cahier des charges des futures sociétés concessionnaires d'autoroutes semblent déjà

L'absence de définition de la location de courte durée dans la loi est très pénalisante quant à la prise en compte de ce service dans l'organisation des politiques de mobilité, et notamment d'électromobilité, alors que ce service est un contributeur clé de la transition écologique des entreprises comme des particuliers. En effet, en l'absence de définition juridique, la location de courte durée n'est pas prise en compte à l'heure actuelle dans les trajectoires de verdissement des flottes d'entreprise, alors même que de très nombreuses entreprises ont recours à des services de location de ce type. Ces services pourraient être intégrés de manière vertueuse dans le verdissement des flottes et dans le des entreprises. De la même manière, la location de courte durée n'étant pas définie, elle n'est pas éligible au forfait mobilités durables qui intègre l'autopartage propre. la location de courte durée est pionnière dans le partage des véhicules : les 250 000 véhicules loués en courte durée sont utilisés par plus de 15 millions d'utilisateurs chaque année. Cette activité de location répond par ailleurs, en tout point, à la définition de l'autopartage faite par le code des transports. Quel est l'avis de la commission

qui provient de la construction du véhicule. Il s'agit d'une pratique vertueuse qui est soutenue par plusieurs dispositifs, notamment le forfait mobilités durables. La location de courte durée s'inscrit dans la même logique, mais n'implique pas nécessairement une réduction du nombre de véhicules du même ordre de grandeur que l'autopartage. de cet amendement conduirait à ce que les autorités organisatrices de la mobilité délivrent des labels d'autopartage à destination de véhicules de location de courte durée,

Je vous remercie, ne soient pas les grands oubliés de la transition écologique, alors même que ce sont ceux pour lesquels l'usage de la voiture s'impose le plus. C'est donc là que les marges de progression sont les plus fortes.

très précis et élaborés du sénateur Jacquin, qui nous ont été remis au début du mois de janvier. Nous avons eu l'occasion d'en reparler en commission. J'ai confié, depuis lors, une mission à Philippe Duron sur ces sujets. Dans un contexte où la crise économique frappe

les outils dont nous disposerons pour faire face de façon conjoncturelle à la crise et, plus systémiquement, pour bien intégrer les territoires les moins denses de notre République à cette réflexion collective. Je demande donc le retrait

est ainsi libellé : La parole est à M. Henri Cabanel. L'article 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite Grenelle 1, dispose qu'afin de rendre plus attractif le transport ferroviaire pour les voyageurs, l'État encouragera le développement du service auto-train. Le service de l'auto-train n'était pas plus onéreux que de prendre dans la voiture tout au long du trajet jusqu'à l'arrivée. Nous le savons, la SNCF a supprimé ce service historique au début de 2020 pour le remplacer par Hiflow, un service de transport routier de véhicules par camion ou par chauffeur. Cela ne constitue certainement pas un progrès environnemental. L'auto-train, considéré comme coûteux, a été abandonné faute de rentabilité, selon la SNCF, à la suite de diminutions de capacités de transport, de réductions de plages horaires et de fréquences. Il y a eu des suppressions progressives de lignes dans l'opacité la plus totale. Pourtant, en 2017, lors du soixantième anniversaire de l'auto-train, la SNCF se réjouissait d'avoir atteint un record historique de 30 % de nouveaux clients. Cet amendement tend à affirmer que l'État s'engage à soutenir le rétablissement et la relance de l'auto-train permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce service public de transport multimodal, qui a toute sa place dans le cadre de la transition écologique.

L'accord de Paris s'applique depuis 2020. Il nous semble donc utile de revenir sur les outils concrets permettant à la France de respecter les engagements qu'elle a contractés pour elle-même. Notre pays peine à atteindre les objectifs de réduction de 27 % de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2028 par rapport à leur niveau de 2013 et de 75 % d'ici à 2050. de l'Observatoire climat-énergie, les objectifs de stratégie nationale bas-carbone n'ont pas été atteints depuis 2016. Le secteur des transports, qui représente environ 30 % de ces émissions, a dépassé de 12,6 % son budget carbone en 2018. On voit donc bien la tendance qui se dessine, celle d'une politique nationale du tout-routier et du tout-aérien, reléguant le ferroviaire au rang de parent pauvre des politiques publiques. Il s'agit pourtant d'un outil écologique, fiable et sûr de maillage des territoires, territoires, apportant une réponse aux besoins de mobilité de nos concitoyens. Dans ce cadre, nous avons déjà exprimé nos préoccupations sur ces questions en organisant un débat sur la relance du service auto-train. Là encore, le scénario est le même, celui du sabotage du service public : en trente ans, le service a perdu 80 % de trafic et les trains auto-couchettes ont totalement disparu, résultat d'une politique coupable de rétraction de l'offre. Les possibilités de substitution promues par l'entreprise, le transport des voitures par camion ou leur acheminement par la route avec un chauffeur, sont un véritable contresens au terme duquel la SNCF devient elle-même pourvoyeuse de solutions routières.

Cet inventaire exhaustif est absolument nécessaire pour que l'État concédant puisse non seulement contrôler la bonne exécution des contrats et les tarifs des péages, mais aussi anticiper au mieux l'état de ces biens à l'expiration des concessions.

En effet, pour que le Gouvernement puisse rendre ce rapport au Parlement, il sera dans l'obligation d'exiger des sociétés concessionnaires un nombre important de documents et d'informations qui mettront en partie en évidence l'état des infrastructures et les travaux réalisés pour assurer leur bon état.

simple état de fonctionnement de la bande de roulement ou prise en compte plus large- couche d'assises, grillage, passage de la faune, imperméabilisation des sols, etc. ? En la matière, en effet, ne pas prendre en compte le bon état de l'ensemble de l'infrastructure serait sans aucun doute une faute à la fois économique, financière et écologique au regard des impacts environnementaux des plus incertains des éventuels travaux qui s'imposeraient et qui seraient forcément émetteurs de gaz à effet de serre et porteurs de nuisances pour la faune, l'environnement et les sols.

à cet objectif en tant que tel, mais je considère qu'il s'agit de le traiter plus directement en faisant respecter les obligations relatives aux biens concédés plutôt qu'en demandant un énième rapport au Gouvernement.

Néanmoins, penser la décarbonation des transports uniquement en termes de réduction des émissions du transport routier ne semble pas suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques. La transformation du transport routier est indispensable, mais elle prendra du temps. Le développement des modes de transport propres comme le ferroviaire ou le fluvial semble indispensable. La commission a d'ailleurs été sensible à cette question en introduisant plusieurs dispositions

j'espère que ce ne sera plus le cas dans quelques années, quand nous aurons atteint nos objectifs pour doubler la part du fluvial et du ferroviaire -, il est important que ce chapitre fasse également référence au transport routier.

sur la question de la suppression du remboursement partiel de la TICPE pour le transport routier de marchandises. Comme vous le savez, le secteur est confronté à d'importantes difficultés liées à ses marges faibles et à la très forte concurrence plus est, il a été mis à l'épreuve pendant la crise sanitaire. Dans ce contexte, la transition énergétique du transport routier de marchandises soulève de nombreuses questions. En effet, 99 % des poids lourds sont motorisés au diesel.

C'est pourquoi la réduction progressive du remboursement partiel de la TICPE d'ici au 1 janvier 2030 ne saurait s'envisager sans une alternative accessible réelle. La commission, en lien avec la commission des finances et la commission des affaires économiques, a donc conditionné cet objectif à la disponibilité et à l'accessibilité d'une offre alternative et abordable au véhicule, introduisant donc une clause de revoyure. Il s'agit d'une position réaliste qui ne s'oppose pas à la logique initiale du projet de loi, mais qui tient compte des réalités. La commission a par ailleurs adopté plusieurs dispositifs visant à accompagner les transporteurs dans leur transition, par exemple le prêt à taux zéro ou le prolongement du suramortissement

devait faire partie intégrante de la transition énergétique du secteur et demandé au Gouvernement de remettre au Parlement une feuille de route présentant une stratégie claire, détaillée et de long terme sur le verdissement des flottes de camions. Il me semble donc que la rédaction de l'article 30 permet de concilier nécessité de transition et réalisme quant aux technologies disponibles.

Vous comprendrez alors aisément que, si la TICPE collectée par l'État et ensuite remboursée ne l'est plus, on anesthésie les capacités d'investissement déjà faibles de ce secteur. Ce serait paradoxal

À ce problème d'investissement privé se greffe naturellement un problème d'investissement public pour proposer un large réseau de stations d'énergies alternatives, lequel n'existe pas aujourd'hui ou est insuffisamment développé. Les professionnels rencontrés m'ont bien fait comprendre qu'ils avaient intégré la nécessité de verdir la flotte. Essayons toutefois d'être un peu cohérents dans nos approches économiques et, surtout, en

personnellement, je défends le ferroviaire et le fluvial, je reconnais que le transport routier maille le territoire et assure la desserte de l'ensemble

Cela implique de renforcer en amont la sécurité et la traçabilité du transport maritime de marchandises, de responsabiliser les pertes et de clarifier l'information sur le transport de marchandises dangereuses. Les conteneurs, véritables véhicules de la mondialisation, transportent de tout : des produits manufacturés que nous recevons et dont nous avons absolument besoin, des matières premières, des marchandises, même des déchets et des substances dangereuses.

à une simple phrase à visée déclaratoire avec pour horizon 2030. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à prévoir d'ores et déjà une évolution de la fiscalité, puisque celle-ci contribue très clairement à la concurrence déloyale de la route face au rail. Pour autant, un amendement a déjà été adopté en commission pondérant l'objectif d'une flotte plus verte à des « conditions économiques soutenables soutenables ». Cette formulation me paraît assez étonnante, puisque nous pourrons toujours considérer que les conditions économiques ne sont pas réunies : il s'agit en fait de sommes considérables consacrées à chaque loi de finances, cet avantage pesant 1,2 milliard d'euros chaque année. Je souligne que les sommes avancées pour le rail sont assez faibles et pas du tout en rapport avec ce que coûterait la régénération du rail, particulier le soutien au fret qui fera sûrement l'objet d'autres débats. En résumé, nous estimons que cette réserve tue dans l'oeuf toute volonté de réduction des avantages fiscaux pour la route. C'est pourquoi nous revenons à la rédaction initiale, qui était

Si l'on veut accélérer la décarbonation du transport de marchandises, que ce soit par le report modal, l'optimisation de la logistique et le verdissement des flottes de poids lourds, on a besoin de se servir du levier de l'incitation fiscale. souligné, l'article 30 aligne la fiscalité du gazole des transporteurs routiers sur la fiscalité du gazole des automobilistes d'ici à 2030. L'objectif est le bon,

avec la commission des finances et la commission des affaires économiques, a proposé de conditionner la suppression de l'avantage fiscal à l'existence d'une offre alternative et abordable de poids lourds décarbonés. a l'apparence du bon sens, mais elle risque fort d'inciter à l'inaction, alors même que les gains de cette fiscalité seront nécessaires pour investir à la hauteur dans le développement de l'offre de poids lourds moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins polluants.

de maintenir une chaîne logistique, d'assurer un approvisionnement de nos usines, de nos commerces, des villes et des villages français. Le transport routier de marchandises représente 89 % des flux de marchandises et 6 % du total des émissions de gaz à effet de serre.

à l'horizon de 2030, qui représente environ 1,2 à 1,3 milliard d'euros, ne ferait que ralentir les investissements des entreprises en faveur de cette transition énergétique. Cet amendement vise donc à fixer la fin de la fiscalité relative au gazole professionnel au 1 janvier 2040 plutôt qu'au 1 janvier 2030. 2030. Cela permettrait une adéquation avec la mise sur le marché de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative et du réseau d'avitaillement correspondant. Cela permettrait aussi une mise en cohérence

Si on voulait limiter les émissions de CO2 en tuant purement et simplement nos acteurs économiques, on ne s'y prendrait pas autrement ! La France risque ainsi

Cet amendement a pour objet de fixer la date de fin du remboursement partiel de la TICPE sur le gazole professionnel à 2035. Il est en effet difficilement concevable d'arrêter totalement la vente de véhicules de transport routier de marchandises principalement à énergie fossile plus tôt.

hydrogène n'est pas encore décarbonée et mature. Ainsi, les motorisations alternatives ne sont pas encore sur le marché. Il est impératif de tenir compte de l'ensemble de ces éléments,

L'article 30 fixe une trajectoire de réduction de l'avantage fiscal dont bénéficient les poids lourds du transport routier de marchandises sur le gazole jusqu'à sa suppression au 1 janvier 2030. la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à conditionner la suppression de l'avantage fiscal sur la TICPE du transport routier de marchandises à l'existence et à la disponibilité d'une offre alternative abordable. Nous nous opposons à l'intégration d'une telle clause, qui risquerait, d'une part, de repousser la fin de l'avantage fiscal dont bénéficient les poids lourds et, d'autre part, de réduire les efforts et les innovations en matière d'offre alternative de véhicules bas-carbone

Nous souhaitons le rappeler, la révision à la hausse de la TICPE proposée par la Convention citoyenne pour le climat vise à rééquilibrer les coûts avec le fret ferroviaire. Sur l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement à fixer à la France l'objectif de doubler les parts modales de fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici à 2030. Pour atteindre de tels objectifs, le développement du transport combiné rail-route, dans une logique de complémentarité des modes,

le recours aux biocarburants. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur le sujet, mais la répétition n'est pas inutile. Tous les biocarburants n'ont pas un bilan carbone positif. Leur production peut également consommer beaucoup d'énergie et dégrader leur bilan énergétique. Pour ces raisons, nous estimons nécessaire de préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique. Notre objectif est donc double : renforcer le soutien au transport combiné et orienter les aides vers les biocarburants durables.

nous considérons utile de préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé soit vers les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique, soit vers les biocarburants durables.

n'est pas disponible ou accessible en 2030, l'objectif devra être revu. C'est le sens de la clause de revoyure.

de début de la trajectoire de réduction de l'avantage fiscal sur la TICPE. De telles propositions semblent assez peu réalistes, compte tenu de l'absence d'offre de « poids lourds propres » sur le marché. Leur mise en oeuvre

de préciser que les biocarburants utilisés pour la transition énergétique du transport routier de marchandises sont ceux qui présentent un bilan énergétique vertueux.

pays ne pourra pas tenir l'engagement que nous avons voté au début de l'examen de ce texte sans une stratégie rapide sur le transport routier. C'est une évidence absolue. sommes dans l'obligation d'avoir une stratégie volontariste dans les dix prochaines années. Je le rappelle, la lutte contre le dérèglement climatique se joue non pas en 2040, mais bien plus en 2030.

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s'inscrit pleinement dans le cadre de l'économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires. Celui dont je parle est produit localement et ne confisque pas non plus de terres agricoles. En outre, il peut être utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.

Comme un tel biocarburant, même intégré à hauteur de 60 % dans un diesel classique, offre des réponses aux enjeux du développement durable et de l'économie circulaire, nous proposons d'étendre aux esters méthyliques d'acides gras en B60 les allégements de TICPE aujourd'hui réservés aux seuls biocarburants B100, tout en fixant

un effet d'aubaine pour le B60 alors que ce dernier est par définition plus émetteur de gaz à effet de serre que le B100- cela a été souligné -, puisque l'incorporation

Comme cela a été dit à plusieurs reprises depuis le début de nos travaux, la pollution de l'air tue. Elle coûte cher à nos concitoyens et leur prend leur santé. En la matière, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 24 octobre 2019, un arrêt contre la France. Elle a constaté que notre pays n'avait pas respecté les valeurs limites applicables aux concentrations de dioxyde d'azote dans douze agglomérations et zones de qualité de l'air, et qu'il n'avait pas veillé à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, comme l'exige la directive 2008/50/CE.

éviter les sanctions, la France doit agir fortement et ne pas se contenter de renvoyer à 2030 la fin hypothétique des exonérations fiscales sur le transport routier.

pour engager la nécessaire transition vers des transports plus soutenables comme le transport ferroviaire ou le transport fluvial. Ce relèvement de la TICPE pour le transport routier de marchandises, qui figurait

Je ne vous rappellerai pas l'état déplorable de nos ponts, comme l'a montré un excellent rapport sénatorial, ou encore celui de certaines lignes de train. Nous ne proposons pas le transfert de ces infrastructures aux collectivités, mais bien le retour d'un État stratège dans le cadre d'une politique d'aménagement ambitieuse.

sur le secteur des poids lourds, et c'est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à accélérer le verdissement des flottes et à créer une écotaxe assortie d'une suppression de la taxe à l'essieu et d'une bonification du remboursement des taxes sur les carburants. Nous tenons par ailleurs à souligner que le secteur privé a bénéficié,

Nous proposons de relever progressivement dès 2023 la taxation du gazole des transporteurs routiers pour la rapprocher chaque année un peu plus de la fiscalité du gazole des automobilistes. Les gains de cette modification de la fiscalité pourraient évidemment servir au soutien et à l'accompagnement renforcé des professionnels du secteur du transport routier de marchandises pour les aider dans cette transition.

Au regard de ce problème, le maintien de l'exonération de la TICPE pour les navires, qui coûte chaque année 697 millions d'euros à l'État, est difficilement justifiable. Cette exonération a déjà été supprimée pour les engins du BTP en 2020. Dans un souci de cohérence, cet amendement tend à mettre fin à cette exonération pour les navires d'ici à 2030, en commençant dès 2023. L'État pourra ainsi réinvestir ces sommes dans la transition.

Mme Catherine Belrhiti. L'article 30 vise à favoriser la prise en compte du fret ferroviaire au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le transport par fret ferroviaire apparaît crucial pour le bilan carbone régional et national. Un train de marchandises émet quatorze fois moins de CO2 par kilomètre qu'un poids lourd pour une masse transportée équivalente. Une tonne de marchandises transportée par le rail nécessite six fois moins d'énergie et émet neuf fois moins de CO2 que lorsqu'elle Un train de fret transporte plus de 500 tonnes de marchandises, soit l'équivalent d'une trentaine de camions sur la route. Le fret ferroviaire n'a donc que des vertus écologiques. La France compte 30 000 kilomètres de voies ferrées, dont 2 800 kilomètres de lignes à grande vitesse (LGV).

projet de loi prévoit son doublement à l'horizon de 2030. Il faut donc promouvoir le fret ferroviaire et tout mettre en oeuvre pour une transition du transport routier vers le transport par train.

Dès lors, conformément à l'article 47 de la directive 2012/34/UE, le présent amendement vise à identifier les sillons sur lesquels les trains de fret pourraient circuler la nuit sur toutes les lignes, y compris à grande vitesse. C'est la mission que cet amendement entend confier au Sraddet.

à faire du fret ferroviaire une priorité, notamment la nuit, mais l'identification des lignes dédiées dans le Sraddet n'est peut-être pas le moyen le plus opportun pour y parvenir. Je sollicite l'avis du Gouvernement.

Ils souhaitent par ailleurs que le rapport annuel que le Gouvernement devra transmettre au Parlement détaille les mesures prises pour favoriser le report modal et encourager l'intermodalité, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette stratégie. Quel

tout en limitant le recours aux transports routiers terrestres. Nous avons tous à y gagner : massification du transport de marchandises, amélioration de la qualité de l'air dans les grandes zones urbaines, qualité de vie, développement de nos ports, à l'heure où le futur canal Seine-Nord constituera un levier de développement économique important. Quel est l'avis de la commission ? Doubler la part

de doublement de la part du fret ferroviaire d'ici à 2030. Nous pensons d'ailleurs que cet objectif pourrait être complété par celui de 25 % de l'ensemble du transport de marchandises d'ici à 2050, fixant ainsi un cap clair. Cette ambition a toutefois besoin de moyens. Nous avons formulé au travers de nos amendements un certain nombre de pistes, notamment celle de l'écocontribution sur les billets d'avion, qui permettrait d'engranger 4,2 milliards d'euros, de quoi financer notamment la remise à niveau des infrastructures. Cette Cette ambition a aussi besoin d'outils, et Fret SNCF en est un. L'État, actionnaire unique de la SNCF, doit jouer son rôle d'aménageur au service de la transition écologique. Nous avons déposé une

enfermé dans une logique comptable. Il doit bénéficier de moyens financiers, matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de son rôle de service public au service de la Nation. Nous proposions même

J'ai parlé un peu plus tôt des soutiens au secteur du transport combiné, du wagon isolé et de la réouverture d'un certain nombre d'autoroutes ferroviaires pour être au rendez-vous du report modal. Ce sont autant d'éléments qui forment un socle très solide pour dynamiser le fret ferroviaire dans notre pays.

Hervé Maurey, visent à compléter l'article 30 du présent projet de loi, qui prévoit, sur l'initiative du rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, un objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici à 2030. L'amendement n° 1059 rectifié prévoit que la stratégie gouvernementale pour le développement du fret ferroviaire et du transport fluvial soit assortie d'une programmation financière pluriannuelle. Quant à l'amendement n° 1060 rectifié, il vise à ce que le Gouvernement, dans sa stratégie relative au fret ferroviaire, donne de la visibilité sur le système d'aides

et de marchandises, mais il ne me semble pas pertinent d'ajouter cet item parmi la liste des indicateurs de suivi de la stratégie nationale de développement des modes massifiés, dans la mesure où l'électrification à quai n'a pas de lien direct avec le développement des modes ferroviaires et fluviaux. En conséquence, l'avis est défavorable. Quel est

marque de relance du fret ferroviaire et de sa pertinence pour les entreprises. La question de l'utilisation de ces installations est également importante : de nombreux sites sont raccordés en théorie, mais beaucoup d'installations sont en réalité dormantes. En 2019, le Cerema notait que 62 % des ITE ne recevaient pas de trains de marchandises.

article inscrit dans la loi l'objectif du doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial d'ici à 2030. Il définit également « une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés

Si le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain se félicite de l'adoption, par la commission, de cette disposition, alors que le Gouvernement tarde à rendre publique cette stratégie, dont la publication était pourtant prévue, en vertu de la LOM, pour le 1 janvier 2021

Il s'agit par exemple de l'organisation industrielle dans les territoires ou du type de biens à transporter, des niveaux de services exigés par les commanditaires de service de transport- flexibilité, coût logistique total -ou bien de la compétition avec le transport routier sur un ensemble de flux.

les industriels- chargeurs ou logisticiens -et les gestionnaires de flux. Ces informations sont très importantes pour les pouvoirs publics, pour le gestionnaire d'infrastructure et pour les opérateurs ferroviaires chargés des investissements et de la rentabilisation de ces lignes.